La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 10 octobre 2019 a été publié sur le site internet du Sénat.

de l'économie et des finances. Ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé. L'accès aux soins et aux services de santé est la préoccupation majeure des Français. La désertification médicale touche une grande partie de la France des campagnes et des petites villes. Elle menace de virer à la crise sanitaire si des solutions innovantes, simples et efficaces ne sont pas mises en place rapidement. Supprimer le est une décision salutaire, mais partielle. En 2025, la France atteindra le pic bas du nombre de médecins en exercice. Dans cette perspective, il faut agir sans tarder Ainsi, parmi les solutions à disposition, je veux mettre en lumière le dispositif PAIS, plateforme alternative d'innovation en santé. Imaginé et développé dans mon canton du département de Loir-et-Cher par un médecin hospitalier et un directeur d'hôpital, il propose aux médecins généralistes une forme d'organisation alternative, plus souple et plus adaptée aux nouvelles attentes et pratiques des médecins généralistes de proximité. revitalise l'offre de médecine de proximité en favorisant les synergies entre médecins, au sein d'un même bassin de vie. Cela passe, par exemple, par la mutualisation du secrétariat, afin de filtrer les appels et alléger les tâches administratives, et par l'organisation à tour de rôle de la prise en charge des soins sans rendez-vous. En Loir-et-Cher, les résultats sont là : amélioration des conditions de travail des médecins, meilleur accès aux soins de proximité et réduction du recours aux urgences hospitalières et aux sapeurs-pompiers. PAIS, une nouvelle médecine de proximité est possible. C'est une réponse innovante et pertinente à la question de la démographie médicale et à l'équilibre géographique de l'offre de soins. Gouvernement est-il disposé, avec l'appui des médecins qui le souhaitent, à généraliser ce dispositif à l'échelle nationale et, si oui, à quelle échéance ? La

la question qui a été transmise au ministère de l'économie et des finances et à laquelle je devais vous apporter une réponse ce matin concernait la labellisation du secteur de la pâtisserie,

Bien évidemment, je lui transmettrai cet élément d'information et vous savez l'intérêt qu'elle porte au développement de solutions alternatives, différentes et innovantes pour préserver la présence médicale dans les territoires.

et vous avez souligné combien le dispositif mis en place dans votre département permettait d'atteindre cet objectif -, tout en préservant un accueil médical de qualité sur tout le territoire, quelles que soient les formules retenues. Se posera ensuite la question

les possibilités d'accès aux études de médecine permettra d'avoir des médecins après plusieurs années de formation. Nous avons donc encore quelques années difficiles devant nous en matière de démographie médicale. C'est aussi la raison pour laquelle, au-delà des présences médicales sur le territoire que vous avez évoquées, s'exprime la volonté d'organiser différemment les soins, par exemple en permettant à des infirmiers de pratiquer un certain nombre d'actes de manière à rendre plus efficace l'accueil des patients. le dispositif que vous présentez a intéressé Agnès Buzyn, qui vous a dit son souhait d'en savoir plus : je lui transmettrai votre question et je ne doute pas qu'elle reviendra vers vous pour en prendre connaissance de manière plus précise, voire, si vous lui en faites l'invitation, pour le découvrir sur place.

Avant 2017, les valeurs locatives étaient établies en référence à des données datant de 1961 pour les propriétés non bâties et de 1970 pour le foncier bâti. Cette méthode ne reflétant plus la réalité du marché, des travaux de révision des valeurs locatives étaient nécessaires. Ils ont débuté à l'échelon départemental en 2010 pour s'achever en 2017. Ainsi, depuis le 1 janvier 2017, tous les locaux professionnels entrant dans le champ de la révision disposent d'une nouvelle valeur locative révisée, égale au produit de la surface pondérée par un tarif au mètre carré, éventuellement ajusté d'un coefficient de localisation. Le secteur de l'hôtellerie de plein air est visé par cette révision les valeurs locatives des locaux professionnels sont dorénavant assises sur des valeurs calculées à partir des loyers réels constatés. Le degré d'augmentation de cette taxe n'était pas connu et il apparaît que ces nouvelles classifications ont entraîné de grandes disparités entre les départements et relevé certaines valeurs locatives à des taux excessivement élevés, notamment dans mon département du Var. L'hôtellerie de plein air a un poids économique important au sein de ce département, qui se classe parmi les premières destinations touristiques françaises. Le Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var, qui regroupe 180 campings adhérents, compte 1 574 équivalents temps plein salariés, soit 64 millions d'euros de salaires versés annuellement. Mon département est très touché par les conséquences disproportionnées de cette révision. Une nouvelle révision plus appropriée est réclamée par le Syndicat de l'hôtellerie de plein air, car, avant la réforme, l'évaluation et les critères pris en compte aboutissaient à un prix du mètre carré compris

plus de dix fois dans 42 % des cas, entre cinq et dix fois dans 32 % des cas. Dans ces conditions, je demande à M. le ministre une réévaluation des valeurs locatives pour prendre en compte la situation spécifique du secteur de l'hôtellerie de plein air et appliquer un niveau de taxation adapté et, surtout, conforme aux dispositions prises dans les départements voisins. Je souhaite également que soit organisée une table ronde avec l'ensemble des acteurs institutionnels, afin de trouver des solutions durables et de travailler en parfaite transparence avec les services fiscaux du Var. La parole

La valeur locative est déterminée à partir de données individuelles du local professionnel, comme la surface principale et secondaire ou encore la catégorie d'imposition, et de paramètres départementaux, comme le secteur locatif, le tarif au mètre carré ou encore le coefficient de localisation. Tous ces paramètres ont été validés au plus près du terrain par des commissions départementales réunissant des représentants des entreprises et des collectivités territoriales. Afin de limiter les fortes variations à la hausse comme à la baisse par rapport à l'ancien système d'évaluation, la mise en oeuvre de la révision au 1 janvier 2017 s'est accompagnée de dispositifs atténuateurs sur la valeur locative et la cotisation de taxe foncière pour rendre soutenable la réforme, avec un dispositif de planchonnement et de plafonnement, de telle manière que les convergences, s'il y a lieu, puissent prendre le temps nécessaire. Cela étant, pour tenir compte des fortes augmentations de taxe foncière de certains établissements de plein air, situation que vous avez soulignée, les services de la direction générale des finances publiques mènent actuellement un travail d'analyse afin de s'assurer de la correcte évaluation des établissements concernés. En effet, comme vous, nous avons pu constater un certain nombre de variations extrêmement importantes. Cette démarche est en cours : elle est partagée avec la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et elle nous semble de nature à répondre aux préoccupations que vous avez exprimées. Ce travail de clarification, qui est assez technique, prend du temps et nécessite et nécessite aussi une clarification doctrinale en matière d'établissements en plein air, sera poursuivi dès l'année prochaine par les travaux de mise à jour des secteurs locatifs et des tarifs prévus à l'article 1518 du code général des impôts. Je pense que les travaux que les travaux menés à la fois sur un plan doctrinal, sur un plan d'évaluation et pour modifier l'article 1518 du code général des impôts permettront d'apporter une réponse satisfaisante à la question que vous avez posée et aux préoccupations que vous avez relayées.

Ne pouvant entrer dans le champ d'application de l'article 1382 du code général des impôts, les musées détenus par des associations sont pleinement soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette imposition constitue une indéniable charge pour les associations propriétaires et met en péril leur avenir. Cette situation interpelle particulièrement, puisqu'elle vient pénaliser des activités à but non lucratif, qui reposent sur le bénévolat et dont la portée est d'intérêt général.

village de 140 habitants. Elle les a restaurées, puis aménagées en un écomusée, qui met aujourd'hui en valeur l'histoire, les traditions et le patrimoine de l'ancienne cité fortifiée de Châtillon-sur-Saône. Reposant sur le seul dévouement des bénévoles, ce musée ne dispose pas des moyens suffisants pour équiper les locaux de toilettes ou d'évacuation d'eau. Les recettes des entrées ne couvrent pas davantage les frais d'entretien et de gardiennage. Seules les fêtes et les animations de rue organisées tout au long de l'année par les bénévoles

l'avenir est, de la même manière, remis en cause. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, au regard du rôle majeur que ces associations jouent en faveur de la préservation du patrimoine et de l'accès du plus grand nombre à la culture, je souhaiterais savoir si un aménagement fiscal était envisageable pour répondre à ces difficultés.

à la taxe foncière sur les propriétés bâties des associations à but non lucratif propriétaires de musée. Plus spécifiquement, puisque vous avez conclu par cette question, vous souhaitez savoir si le Gouvernement envisage de leur accorder un abattement ou une exonération applicable aux propriétés publiques. Comme vous le savez, la taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt réel dû à raison de la détention d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite ou les revenus du propriétaire. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent rester une exception- c'est la doctrine constante que nous observons. Par ailleurs, je souligne que, si les immeubles qui appartiennent à l'État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics d'assistance scientifique ou d'enseignement sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est à la double condition d'être affectés à une mission de service public et d'être improductifs de revenus pour le propriétaire des bâtiments. Ce sont ces sujétions qui justifient la différence de traitement entre établissements publics et privés, quand bien même, vous l'avez souligné, les revenus tirés de ces bâtiments restent modestes, ne suffisant pas forcément à faire face à un certain nombre de charges. En outre, si nous accédions à cette demande, des mesures similaires pourraient être sollicitées par d'autres structures associatives d'utilité générale, certainement tout aussi dignes d'intérêt, sans que nous puissions en maîtriser les impacts budgétaires. Enfin, un tel allégement fiscal induirait une perte de ressources pour les collectivités territoriales, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. C'est la question que nous devons nous poser chaque fois qu'une exonération de fiscalité locale est accordée. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'est pas favorable à l'aménagement que vous appelez de vos voeux. Je précise cependant

mais aussi coût pour les collectivités qui les financent. C'est pourquoi je souhaite vous interpeller sur un sujet peut-être technique, mais pourtant très important : la tarification et la comptabilité des Ehpad. En effet, les conseils départementaux sont chargés d'établir chaque année la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) habilités à l'aide sociale. dans ce cadre, des investissements importants, sur un projet de réhabilitation, peuvent avoir un impact important sur le prix de journée- de l'ordre de 15 à 20 euros quelquefois -, ce qui est difficilement supportable par les familles. Afin d'anticiper et de lisser une telle augmentation, il serait pertinent pertinent de pouvoir provisionner l'impact de ces évolutions tarifaires. Cela est possible pour les établissements soumis à la nomenclature comptable M22, mais pas pour les Ehpad, soumis à la nomenclature comptable M21.

en autorisant, comme pour la M22, la constitution de provisions dédiées au projet immobilier de l'établissement ? La parole est à M. le

Voici les précisions que je puis apporter à votre question. Ces établissements sont financés par l'assurance maladie au titre des prestations de soins, par le département au titre des prestations afférentes à la dépendance et par l'usager au titre de l'hébergement ou par le département lorsque ce résident bénéficie de l'aide sociale à l'hébergement. Pour accueillir ces bénéficiaires, les Ehpad sont alors habilités par le département et le tarif afférent à l'hébergement est fixé par le président du conseil départemental ; il est déterminé en fonction des charges prévisionnelles de l'établissement. Or, lorsqu'un Ehpad réalise d'importants travaux de réhabilitation- vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur -, de nouvelles charges sont générées par les immobilisations issues de ces travaux, notamment en matière d'amortissement, et par d'éventuels frais financiers liés à la souscription d'emprunts. Ces charges d'amortissement et financières peuvent conduire à augmenter, à due concurrence, le prix de journée lié à l'hébergement en Ehpad. Afin de limiter la hausse des tarifs d'hébergement et le reste à charge que les investissements induisent pour les résidents, les arrêtés des 10 novembre 2008 et 16 juin 2014 relatifs aux instructions budgétaires et comptables M22 et M21 prévoient que les autorités de tarification peuvent verser aux Ehpad une allocation anticipée destinée à compenser les charges d'amortissement et les frais, financiers ou non, liés à des opérations de rénovation ; ces crédits font l'objet d'une provision réglementée pour renouvellement des immobilisations.

À cet effet, les instructions M21 et M22 prévoient un compte de provision réglementée pour renouvellement des immobilisations. Enfin, les Ehpad ont également la possibilité, dans le respect des dispositions prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé avec les autorités de tarification compétentes, d'affecter un résultat d'exploitation excédentaire

pour compenser les charges d'amortissement induites par les nouveaux équipements de mise aux normes de sécurité. De même, cette réserve de compensation peut être constituée par l'ensemble des Ehpad publics, qu'ils relèvent des instructions M21 ou M22. Aussi les instructions M21 et M22 offrent-elles les mêmes possibilités aux Ehpad en matière de provisionnement et de financement des charges liées à des investissements. Cette analyse du ministère de l'action et des comptes publics est partagée par la direction générale de la cohésion sociale.

des comptes publics. Monsieur le secrétaire d'État, le projet du Gouvernement pour les Hauts-de-Seine est de fermer l'intégralité des 19 trésoreries municipales, la moitié des 16 services des impôts pour les particuliers et les trois quarts des services des impôts pour les entreprises. Ce plan de destruction du service public a été décidé sans aucune concertation avec les salariés et encore moins avec les collectivités territoriales. Dans un geste d'une grande clémence, vous avez décidé d'arrêter le bras du bourreau pour l'année 2020. Est-ce à dire, monsieur le secrétaire d'État, que toutes ces suppressions interviendront en 2021 ? Par ailleurs, votre gouvernement a annoncé que les buralistes et la Française des jeux, bientôt privatisée, seront habilités à recevoir le paiement des impôts. C'est le retour de la ferme générale organisée par Colbert en 1680. Du haut de ce plateau, il doit sourire devant la fulgurante nouveauté de ce retour en arrière prodigieux

il se trouve que le réseau des finances publiques a connu des centaines de fermetures depuis la fin des années 1990. Nous parlons de 1 200 fermetures depuis 2000, avec un rythme, sur dix ans, d'environ 120 fermetures par an. Ces fermetures ont été décidées dans le cadre de plans annuels de restructurations de services, qui ne tenaient bien souvent pas compte des engagements pris l'année précédente auprès des maires ou des collectivités. Gérald Darmanin et moi-même avons voulu changer cette méthode et nous souhaitons travailler de manière pluriannuelle, avec quatre objectifs : premièrement, augmenter le nombre d'accueils de proximité en association avec les préfets, en concertation avec les élus et en lien avec l'évolution d'autres points d'accueil du service public, comme les maisons France services ; deuxièmement, répondre de manière plus satisfaisante au besoin de conseil des élus locaux en dédiant 1 200 cadres à cette mission de conseil financier partout sur le territoire, en veillant à ce que chaque maire membre d'une même intercommunalité ait le même conseiller financier ; troisièmement, créer des équipes de travail plus étoffées avec une organisation plus satisfaisante, car, dans bien des départements- ce n'est pas nécessairement le cas des Hauts-de-Seine -, les équipes sont désormais trop petites en taille et trop réduites en nombre pour offrir un cadre satisfaisant aux agents publics ;

Le projet a été présenté au mois de juin dernier à l'Association des maires des Hauts-de-Seine, puis aux parlementaires du département et à chaque maire concerné. Il prévoit la création de postes de conseillers auprès des décideurs locaux, comme c'est le cas dans tous les projets départementaux. Il prévoit aussi de mieux prendre en compte la montée en puissance et l'affirmation des établissements publics territoriaux en créant un service de gestion comptable pour chacun des quatre territoires du département. Nous précisons aussi qu'un regroupement des services de gestion permettra de disposer de services de plus grande taille, mieux à même de traiter un certain nombre de tâches. La concertation va se poursuivre autour de ce projet pour faire en sorte qu'il soit le plus partagé et le plus adéquat possible avec les besoins du territoire. Il doit aussi tenir compte de la fréquentation par le public d'un certain nombre de points de contact des finances publiques. En effet, du fait des réformes fiscales qui sont menées et de la dématérialisation, la fréquentation est beaucoup moins importante.

montant et de manière totalement anonyme et confidentielle, sans que l'origine du paiement puisse être retracée, des sommes qu'ils doivent au Trésor public, aux heures d'ouverture des buralistes, lesquelles sont, vous en conviendrez, souvent plus en adéquation avec les rythmes de travail de nos concitoyens.

de l'Europe et des affaires étrangères. J'appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la contestation de la souveraineté de la France sur le Tombeau des rois par des rabbins israéliens issus de la mouvance ultra-orthodoxe. Le Tombeau des rois, situé à Jérusalem-Est dans la partie palestinienne de la ville annexée en 1967 par Israël, appartient au domaine national français en Terre sainte depuis la fin du XIX siècle. Le Hekdesh du Tombeau des rois, association cultuelle juive, a engagé le 15 mai 2019 une procédure judiciaire en France son défenseur, en assignant le ministère des affaires étrangères et le consulat de France à Jérusalem devant le tribunal de grande instance de Paris. Les plaignants revendiquent la propriété du monument, qui constitue le plus grand complexe funéraire de la région. Deux fois millénaire, le Tombeau des rois a été récemment restauré par la France. Cette procédure judiciaire engagée contre l'État français, qui met en cause la propriété française d'un monument situé dans le quartier musulman de Cheikh Jarrah, fait partie d'une stratégie globale de « grignotage territorial » de la part des nationalistes religieux. Aussi, je souhaite que le ministre puisse rappeler solennellement les droits de la France sur le site du Tombeau des rois à Jérusalem.

de la France. Permettez-moi tout d'abord de revenir, comme vous l'avez fait, sur l'histoire et le statut du Tombeau des rois et d'en rappeler l'importance. Il s'agit d'un site archéologique datant du I siècle avant Jésus-Christ, situé à Jérusalem-Est, à quelques centaines de mètres de la vieille ville. C'est donc l'un des rares vestiges antérieurs à la destruction de la ville par Hadrien, en 135 de notre ère. Il a fait l'objet de fouilles par des archéologues français dès les années 1860 avec, à l'époque, la permission des autorités ottomanes. Il s'agit de l'un des quatre domaines nationaux français de Jérusalem, avec l'église Sainte-Anne, le site de l'Eléona sur le mont des Oliviers et le couvent d'Abou Gosh. Le site du Tombeau des rois a été légué en 1886 à la France par les frères Pereire. La République française, représentée par le consulat général de France à Jérusalem, est depuis cette date l'unique propriétaire du site. Aussi, nous ferons valoir notre titre de propriété, également reconnu à l'échelon international par l'accord de Constantinople, dans le cadre des procédures qui seraient engagées. En outre, en tant que propriétaire et seul responsable de la gestion du site, la France a conduit d'importants travaux de sécurisation, de restauration et d'aménagement, afin que le Tombeau des rois- comme les autres domaines nationaux français à Jérusalem -reste accessible à un public varié et selon des modalités adaptées à la préservation et à la dignité des lieux, ainsi qu'à la sécurité des visiteurs. C'est donc véritablement à regret que de violents incidents survenus à la suite de la réouverture du domaine public, le 27 juin dernier, nous ont contraints à procéder à la suspension temporaire de ces visites. Alors que les individus qui ont semé le trouble devraient dire merci à la France d'avoir restauré ce domaine et fait en sorte qu'il demeure un joyau,

Notre secrétaire général s'en est ouvert à l'ambassadrice israélienne avec une note verbale invitant une nouvelle fois Israël à s'exprimer sur la question du droit de propriété. Je le répète, il n'y a aucune ambiguïté en droit comme dans la réalité : la France est propriétaire de ce site.

Je ne reviens pas sur le diagnostic lié à la multiplication de ces meublés de tourisme avec la montée en puissance des plateformes numériques spécialisées.

un numéro d'enregistrement peut être instauré dans un certain nombre de territoires et, dans les territoires qui ne sont pas visés, par décision du préfet sur proposition du maire par le biais d'une procédure sur laquelle je ne reviens pas. Dans la pratique, la loi concernant la déclaration simple d'une mise en location en mairie n'est pas respectée, notamment parce que les hébergeurs ne se déclarent pas toujours en mairie, de sorte que les offices de tourisme ou les mairies n'ont pas de visibilité sur le parc de logements saisonniers. À titre d'exemple, dans une intercommunalité tarnaise, après un petit tour sur les réseaux sociaux, il apparaît qu'à peu près la moitié des meublés de tourisme sont effectivement déclarés. En outre, la pratique de ce numéro d'enregistrement est différente suivant les préfectures. Ma question concerne donc les conditions dans lesquelles les préfets

comment harmoniser les choses et faire en sorte que ces numéros d'enregistrement et la connaissance par les communes des meublés de tourisme puissent être sensiblement améliorés ? La parole

à la fois les loueurs en meublé et l'action des communes en la matière. En effet, la demande du maire doit reposer sur une analyse de l'existence d'une tension locale sur le marché du logement. C'est pourquoi

Merci

de l'intérieur. Monsieur le secrétaire d'État, les forces de l'ordre organisent régulièrement des évacuations des camps de migrants, notamment dans les communes des côtes de la Manche, notamment à Grande-Synthe. Si l'évacuation de ces camps illicites dans lesquels les populations migrantes survivent dans des conditions sanitaires déplorables ne peut être que saluée, de nombreux retours de ces mêmes migrants sont constatés après chaque opération d'évacuation. La situation du littoral du Nord et du Pas-de-Calais est depuis plusieurs années insupportables, tant pour les maires des communes concernées que pour les habitants de ces territoires, bien sûr. Elle est aussi tragique pour les migrants. Hier encore, deux personnes sont décédées au large des côtes de la Manche. Au-delà des démonstrations de force et des évacuations qui se répètent et se ressemblent, mais n'apportent finalement que peu de solutions pérennes, je souhaite savoir si le Gouvernement compte mener une action plus large s'agissant du suivi des reconduites aux frontières et de l'accompagnement des mineurs isolés.

Très clairement, la région des Hauts-de-France fait face à une pression migratoire particulièrement forte, nous le savons. Vous avez évoqué la dernière opération de démantèlement du campement de Grande-Synthe, le 17 septembre dernier. De telles opérations de démantèlement ont deux objectifs : d'une part, encadrer les flux irréguliers et lutter contre les trafics d'êtres humains ; part, procéder à une mise à l'abri respectueuse des droits fondamentaux de ces populations. Elles nous permettent aussi de connaître la situation administrative de ces personnes

obtenir la délivrance des laissez-passer consulaires (LPC), qui permettent la reconduite aux frontières d'un certain nombre de ces personnes. Le taux de

Devenus les acteurs majeurs du secours aux personnes, les sapeurs-pompiers paient les conséquences de la désertification médicale, du vieillissement de la population, des dysfonctionnements de la régulation médicale ou encore des carences ambulancières. Chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) doivent absorber entre 100 000 et 120 000 interventions nouvelles, au prix d'une mise sous tension croissante des hommes, des matériels et des budgets. Dans mon département, l'Essonne, l'activité des sapeurs-pompiers est très impactée par la situation particulièrement tendue du SAMU 91, qui ne dispose pas des ressources humaines adéquates, notamment d'assistants de régulation médicale, au centre de réception et de régulation des appels. Nos sapeurs-pompiers sont en outre les victimes expiatoires d'une société désinhibée, où la violence frappe tous ceux qui sont détenteurs d'autorité ou porteurs d'un uniforme. J'en veux pour preuve les 57 plaintes déposées par les pompiers depuis le début de l'année dans mon département, dont 4 pour des agressions graves le même week-end le mois dernier. Cette situation ne peut plus durer et nous impose d'agir. Elle vous impose d'agir, monsieur le ministre ! Quelles mesures entendez-vous prendre afin de rendre plus simple, plus rapide et plus efficace la réponse opérationnelle en matière de secours aux personnes ? Les sapeurs-pompiers demandent la généralisation de centres départementaux d'appels d'urgence communs à tous les acteurs- pompiers, police, gendarmerie et SMUR -, avec pour numéro d'appel unique le 112. Accéderez-vous à cette demande ? Par ailleurs, la mobilisation croissante des sapeurs-pompiers pour des missions ne relevant pas de l'urgence vitale met en tension les budgets des SDIS. L'État accompagnera-t-il l'effort financier déjà très important des collectivités territoriales ? Enfin, la violence qui frappe les sapeurs-pompiers, confrontés aux difficultés des cités et à la misère sociale, doit être combattue avec la plus grande énergie.

à six mesures, en cours de réalisation, parmi lesquelles je citerai : la généralisation des coordonnateurs ambulanciers au sein des SAMU-Centre 15 pour diminuer la sollicitation des sapeurs-pompiers pour des missions réalisables par des ambulanciers privés ; la réduction des délais d'attente des sapeurs-pompiers aux services d'urgence afin de limiter les temps d'immobilisation des véhicules de secours et de leurs équipages ; la possibilité pour les SDIS d'effectuer des interventions à deux sapeurs-pompiers, pour

des pompiers. Ce travail complète d'autres initiatives, notamment le projet NexSIS, qui dotera les SDIS d'un outil commun pour mieux gérer les appels et les opérations. Interopérable avec celui du SAMU, de la police nationale et de la gendarmerie nationale,

il appartient de prendre toutes ses responsabilités pour rétablir la confiance avec les soldats du feu. Ils demandent de la considération et un engagement fort des pouvoirs publics dans plusieurs domaines : le secours aux personnes, le volontariat et la sécurité en intervention. La

à l'instabilité juridique liée aux autorisations uniques pluriannuelles délivrées aux organismes uniques de gestion collective de l'eau. Elle concerne également les autorisations de construction de réserves d'eau, toutes attaquées devant les tribunaux, alors que le stockage est l'une des réponses à apporter pour une gestion durable de l'eau. Le tribunal administratif de Poitiers a rendu un jugement le 9 mai annulant les autorisations uniques pluriannuelles sur les bassins de la Charente amont et du Marais poitevin. en résulte l'annulation différée des autorisations administratives de gestion collective de l'eau pour l'agriculture, à compter du 1avril 2021, et une demande de révision des volumes autorisés pour 2019 et 2020. d'une très mauvaise nouvelle, qui met à mal le travail réalisé ces dix dernières années par les organisations agricoles impliquées dans la gestion de l'eau et par les irrigants pour répondre aux nouvelles exigences d'une gestion équilibrée et responsable L'État a fait appel en demandant un sursis à exécution. Peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus, monsieur le secrétaire d'État ? Dans un contexte de changement climatique, les agriculteurs se retrouvent dans une position incertaine pour les années à venir, alors que l'irrigation va devenir une condition pour la pour la production agricole, qu'elle est un facteur de maintien de l'élevage, gage de qualité des produits pour l'aval, vecteur de diversification agricole, favorisant les circuits courts. Les enjeux économiques, sociaux et territoriaux sont particulièrement importants pour nos territoires ruraux. Vous le savez, je l'espère. Monsieur le secrétaire d'État, compte tenu de l'urgence de ce dossier, entendez-vous sécuriser juridiquement les outils de gestion de l'eau et les volumes autorisés pour ne pas déstabiliser les exploitations agricoles et les filières économiques qui s'appuient sur l'irrigation ? La

est essentielle pour l'agriculture. Les conditions extrêmes de cette année nous le rappellent, l'agriculture est l'un des secteurs particulièrement exposés à un risque accru de manque d'eau dans le contexte du changement climatique.

très clairement, irrigation et transition agro-écologique vont de pair. À cet égard, je salue les agriculteurs, qui, en dix ans, ont réduit de 30 % le volume d'eau utilisé pour irriguer leurs cultures. On le voit, cette profession s'adapte

Poitiers. Pour répondre à ces enjeux, faciliter la mobilisation de la ressource et sécuriser les porteurs de projet, le ministère de l'environnement et le ministère de l'agriculture agissent conjointement. Instruction a été donnée aux préfets de faciliter la construction de nouveaux ouvrages dans le cadre de projets de territoire et de donner la possibilité aux agences de l'eau de financer

Le ministre de l'agriculture m'indiquait dans une réponse du 19 juillet qu'il était important d'amplifier la transition agro-écologique afin de maintenir une agriculture riche en biodiversité, respectueuse de la qualité de l'eau et de la richesse de nos territoires. Je souscris totalement

une alerte que le ministère de l'agriculture prend très au sérieux, selon le communiqué officiel. Cette nouvelle progression de met en lumière un problème grave il n'existe aucun traitement curatif efficace, les scientifiques ayant seulement démontré que le réchauffement climatique est un catalyseur et que les insectes de la famille des cigales de cette bactérie. Jusqu'à présent, dans les Alpes-Maritimes, seule la bactérie de souche multiplex avait été décelée sur des oliviers. Pour la première fois, la bactérie de souche pauca, la plus virulente, a été détectée, la même que celle qui décime les oliviers en Italie.

pour l'avenir de leur outil de production puisque, en l'état, l'arrachage obligatoire dans un rayon de 100 mètres autour d'un olivier malade détruit les végétaux sur plus de 3 hectares, ce qui signifie que 300 oliviers sont arrachés et brûlés. Les professionnels ne s'exonèrent pas des mesures nationales de prévention, mais, face à

L'Institut national de recherche agronomique (INRA) a-t-il de nouvelles propositions pour endiguer la progression de la bactérie ? Enfin, une stratégie de lutte à l'échelle européenne devait être mise en place en 2018. Quelles ont été les décisions prises et mises en oeuvre depuis ?

mis provisoirement sous filet anti-insectes et pour évaluer l'intérêt de mettre en place des mesures complémentaires pour une gestion optimale de ces foyers. Nous sommes sensibles aux craintes des producteurs. Depuis 2019, les services du ministère de l'agriculture et de l'alimentation s'appuient sur l'INRA et sur l'Anses pour améliorer les méthodes de surveillance de la bactérie. Les échanges sont permanents entre ces deux structures, très impliquées dans des projets européens, tels les projets XF-Actors et POnTE. À l'échelon européen, la France

dans une lettre de mission datant du 28 mars 2019, quatre ministères mandatent l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales pour mener une mission sur les établissements et services d'aide par le travail (ÉSAT). Au nombre de 1 400, ces établissements accompagnent par le travail 120 000 personnes handicapées. Dans ce courrier, les deux inspections sont missionnées pour interroger le modèle existant et ses principes fondateurs ; répertorier le mode de financement des ÉSAT et leurs liens avec leur environnement, examiner les pistes d'accompagnement vers l'emploi ordinaire ; dessiner des scénarios d'évolution de ces structures. En deux mois, les inspections doivent à la fois remettre des chiffres au Gouvernement et des pistes de scénarios d'évolution des ÉSAT, et ce alors que la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, introduite par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, n'entrera en vigueur que le 1 janvier 2020. De nombreuses associations s'inquiètent de ce calendrier et des intentions du Gouvernement s'agissant de l'évolution des missions

Alors que le rapport était attendu pour le mois de juillet, vous avez souhaité connaître dès le mois de mai les premières pistes d'évolution proposées. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur ces premières propositions ? En signalant, dans un courrier à l'IGAS, que la mission devrait préciser comment mieux répondre à l'objectif d'inclusion et d'individualisation des personnes en situation de handicap, vous souligniez la volonté du Gouvernement de tendre vers une société 100 % inclusive au travers de la « Réponse accompagnée pour tous » (RAPT). À ce jour, le rapport de l'IGAS n'est toujours pas public. Les inquiétudes des personnels des ÉSAT et des entreprises adaptées sont fortes. Madame la secrétaire d'État, allez-vous rendre ce rapport public ? Et si oui, quand ? La loi du 10 février 2005 avait acté l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les ÉSAT et les entreprises adaptées restent des lieux qui ont fait leurs preuves. Supprimer les ÉSAT, ou en réduire de manière significative le nombre, au regard de l'état du marché du travail, serait une grave erreur.

Certaines personnes en situation de handicap peuvent accéder au travail en milieu ordinaire, bien sûr, mais aujourd'hui, le taux de chômage de ces personnes est le double des personnes sans handicap, comme vous l'avez

Je vous remercie le karaté du programme olympique des Jeux de Paris en 2024. L'art martial n'a pas été retenu parmi les quatre sports additionnels proposés que sont le surf, l'escalade, le skateboard et le breakdance. Cette décision est d'autant plus surprenante que la discipline sera présente lors des jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Forte d'une fédération créée en 1975 et comptant plus de 250 000 licenciés inscrits, dans 5 000 clubs, la France a terminé à la première place du championnat d'Europe 2019. Elle a également remporté 38 titres mondiaux, toutes catégories confondues, dont 6 pour l'épreuve par équipe. Le karaté représente un réel potentiel de médailles pour notre pays en 2024. Le dossier présenté respectait en outre les orientations de l'État et les éléments du projet du Comité d'orientation des jeux Olympiques (COJO). Il s'agit d'un sport innovant, à dominante urbaine et ayant un fort impact sur la jeunesse. La décision du CIO constitue une double peine, sachant que les clubs sont représentés en zone urbaine, dans les villes populaires, mais aussi que 120 000 licenciés entrent dans la catégorie des jeunes

Cette nouveauté ajoutée pour les Jeux de Tokyo de 2020 a pour objectif d'aller à la rencontre de nouveaux publics et de renforcer encore plus l'attractivité des Jeux. En juillet 2018, la commission exécutive du CIO a encadré le processus décisionnel pour les nouvelles épreuves des nouveaux sports de Paris 2024. Lors des Jeux de Tokyo de 2020, le quota d'athlètes et le nombre d'épreuves des nouveaux sports étaient prévus en plus du quota de 10 500 athlètes et de 310 épreuves prévus par la Charte olympique. Pour Paris 2024, le CIO a souhaité intégrer le quota d'athlètes et le nombre d'épreuves des nouveaux sports dans ceux qui sont indiqués dans la Charte olympique. L'objectif, vous le savez, est le développement durable. Il s'agit notamment de limiter le coût des Jeux. La proposition du COJO devait donc refléter la vision de Paris 2024. Les Jeux doivent être attractifs pour la jeunesse, innovants, spectaculaires et mettre en valeur des lieux emblématiques français. En accord avec le calendrier établi par le CIO, dix-neuf fédérations internationales, dont la ont été reçues par Paris 2024 entre octobre 2018 et janvier 2019 et ont présenté de solides propositions d'ajouts de nouveaux sports.

inclusifs, praticables hors des stades, et faisant appel à la créativité. Les quatre sports retenus sont le breakdance, l'escalade, le skateboard et le surf. Pour le président du CIO, Thomas Bach, « les quatre sports proposés sont en tous points conformes aux recommandations de l'Agenda olympique 2020. Ils contribuent à rendre le programme des jeux Olympiques plus jeune, plus urbain, avec un meilleur équilibre entre les sexes. Ils offrent la possibilité de se rapprocher de la jeune génération ». Le choix a été extrêmement difficile.

très présent dans les départements ruraux. C'est un sport par excellence, pratiqué par de nombreux jeunes. Les valeurs de ce sport sont fortes et nécessaires, surtout dans la société dans laquelle nous vivons. Être reconnue comme une discipline olympique aurait été un levier puissant et mobilisateur. Nous regrettons que tel ne

et compte tenu des grandes difficultés que connaît le tribunal de grande instance de Laval. Actuellement, la juridiction de Laval compte deux postes non pourvus, deux personnels en arrêt de travail, un mi-temps thérapeutique, sans compter un certain nombre d'arrêts maladie.

Il en est de même pour plusieurs magistrats en arrêt de travail. Ces absences engendrent les difficultés que vous imaginez : audiences annulées, délibérés prorogés, jugements rendus, mais non signés, dossiers clôturés, mais non audiencés, ce qui est préjudiciable aux Mayennais. La situation est telle que le tribunal de grande instance a sollicité l'aide du barreau pour compléter les compositions des juridictions. Le barreau de Laval a répondu favorablement à cette demande, estimant qu'il était de son honneur de venir en aide à sa juridiction. On ne peut que saluer l'esprit de responsabilité des avocats. Il y va aussi bien sûr de l'intérêt des justiciables, qui attendent leur décision et ne comprennent pas la défaillance du service public de la justice. À ces difficultés s'ajoute depuis de nombreuses années le fait que les greffiers et les fonctionnaires de la justice sont en sous-effectifs. En outre, les moyens matériels et informatiques

? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, à titre liminaire, il convient de rappeler que le budget de la justice pour l'année 2019 est en augmentation de 4,5 %. Il s'agit de la deuxième hausse consécutive. Elle traduit une évolution positive des moyens alloués aux juridictions. Cette augmentation, inscrite dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permettra aux juridictions de procéder à différentes évolutions ayant vocation à rendre plus accessible et plus lisible notre organisation juridictionnelle. En recentrant le juge sur son office, les mesures de simplification prévues par la loi contribueront à améliorer le service public de la justice. Par ailleurs, les moyens budgétaires permettront d'allouer de nouveaux emplois aux juridictions. Ainsi, en 2019, 192 postes nouveaux dans les services judiciaires viendront combler pour partie les vacances de postes en juridiction et développer les équipes autour du magistrat. La direction des services judiciaires s'efforce de répartir au mieux les effectifs sur l'ensemble du territoire, tout en tenant compte des spécificités de chaque ressort. S'agissant plus particulièrement des effectifs de magistrats du tribunal de grande instance de Laval, la circulaire de localisation des emplois pour l'année 2019 fixe à 19 le nombre de magistrats nécessaires au fonctionnement de cette juridiction, dont 15 au siège et 4 au parquet. À ce jour, le tribunal ne compte qu'un poste vacant de juge non spécialisé au siège. Au parquet, les effectifs sont au complet. Une attention particulière est portée à la situation globale de la cour d'appel d'Angers. Actuellement, M. le premier président et M. le procureur général disposent respectivement de 5 magistrats placés au siège et de 3 magistrats placés au parquet, qu'ils peuvent déléguer dans les juridictions du ressort pour renforcer leurs effectifs, notamment en cas de congés maladie. Enfin, dans le cadre de la localisation des emplois au titre de l'année 2019 et au regard de l'évaluation de la charge de travail, l'effectif de fonctionnaires du tribunal de grande instance de Laval est fixé à 38 agents. À la date du 15 septembre, 3 postes sont vacants. Ces vacances de poste seront prises en compte dans le cadre des prochaines opérations de mobilité et de recrutement. Par ailleurs, les chefs de cour ont également la possibilité d'affecter des personnels placés du ressort pour résorber, le cas échéant, un stock jugé trop important.

et solidaire. Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur le projet d'implantation d'un parc éolien sur l'estuaire de la Gironde, dit « du Blayais ». Ce projet prévoit l'implantation d'une quarantaine d'éoliennes de 180 mètres chacune par EDF entre Blaye et Mortagne-sur-Gironde.

Elle abrite de nombreuses espèces animales et végétales classées, dont certaines sont en voie de disparition. L'estuaire est aussi un important couloir pour les oiseaux migrateurs, ainsi qu'un espace de repos. L'implantation de ce parc éolien constituerait une menace importante pour la biodiversité de cette zone. Elle pose aussi la question de son futur démantèlement à l'horizon d'une vingtaine d'années. Enfin, la réalisation d'un parc d'éoliennes dans l'estuaire de la Gironde aurait aussi une incidence considérable sur le tourisme fluvial, ainsi que sur l'oeno et l'agro-tourisme. Le développement du projet hydrolien qui figure dans le contrat de partenariat autour du grand port maritime de Bordeaux pourrait être une solution alternative plus respectueuse de l'environnement et de l'économie locale. L'hydrolien présente en outre l'avantage d'avoir un rendement supérieur à celui des éoliennes. Ce projet éolien a déjà suscité de nombreuses oppositions en Gironde et en Charente-Maritime. C'est pourquoi, madame la secrétaire d'État, je souhaiterais savoir quel projet le Gouvernement entend privilégier pour l'estuaire de la Gironde.

n'étant pas stockable, il faut réaliser un maillage territorial auquel la Gironde doit prendre sa part. Le porteur de projet a d'ailleurs engagé une concertation préalable volontaire jusqu'au 12 juillet dernier. Le projet va faire l'objet d'une instruction complète, au même titre que tout projet

discutés, concertés. L'ensemble des politiques de protection de la biodiversité, des paysages et des riverains seront respectées, bien évidemment. Vous mentionnez l'hydrolien.

très élevés. Elle va mettre encore de longues années avant d'être compétitive par rapport à d'autres énergies qui, elles, le sont déjà, comme l'éolien. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement estime qu'il n'est pas opportun d'encourager le développement de cette filière à un stade commercial à court terme

Enfin, nous sommes sur un territoire forestier où nous attachons beaucoup d'importance à la migration des oiseaux. Vous nous dites que la Gironde est peu vertueuse en matière d'énergie renouvelable. Néanmoins, la forêt landaise est un puits de carbone remarquable. Il me semble un peu réducteur de vouloir harmoniser l'installation de l'éolien sans tenir compte des autres ressources du territoire.

sur les problématiques engendrées par la dangerosité pour la santé et l'environnement des terrains synthétiques. Aujourd'hui, la situation reste très préoccupante. Pour rappel, il s'agit de ces milliers d'hectares de gazons artificiels recouverts de granulats de pneus broyés,

En effet, si l'Agence révèle que l'analyse complète des études scientifiques disponibles fait état de faibles risques pour la santé, elle pointe cependant des risques potentiels pour l'environnement et, surtout, des limites méthodologiques rendant nécessaire une analyse plus large et plus approfondie. Il manque une véritable étude épidémiologique à long terme. C'est dans ce contexte que les élus locaux, confrontés à une pression croissante de leurs administrés et faisant face à des dilemmes financiers importants, sont livrés à eux-mêmes pour trancher cette question. Certains choisissent de conclure de très importants marchés publics visant à déposer ces pelouses synthétiques. Cependant, les solutions de recyclage sont loin d'être effectives, ce qui conduit à des situations inquiétantes. Une fois retirées, ces billes de plastique sont soit stockées dans des décharges à ciel ouvert, soit dirigées vers des réseaux de sous-traitance à l'étranger, sans la moindre traçabilité. À l'heure où les scandales industriels mettant en cause la santé de nos concitoyens ou la protection de l'environnement se multiplient, nous devons redoubler de vigilance et ne pas nous éloigner du principe de précaution.

2018, conclut : « les expertises sur les risques liés à l'exposition de sportifs et d'enfants utilisateurs des terrains synthétiques, ainsi que de travailleurs impliqués dans la pose et l'entretien de ces terrains concluent majoritairement à un risque sanitaire négligeable ».

notamment la réalisation d'un guide de bonnes pratiques pour l'installation des terrains synthétiques. C'est à ce titre que le ministère de la transition écologique et solidaire, en collaboration avec le ministère des sports, a engagé la mise en place d'un groupe de travail pour la rédaction de ce guide. Ce groupe associera des professionnels de la fabrication et de l'aménagement des terrains, les collectivités locales et les organisations en charge du recyclage des pneumatiques usagés, en vue d'avancer collectivement à l'élaboration de ce guide de bonnes pratiques.

dans les granulats, selon le principe de précaution. La Commission devrait soumettre rapidement cette mesure au vote des États membres. Par ailleurs, un projet de renforcement de la réglementation pour interdire les microplastiques est en cours d'expertise technique par l'Agence européenne. Il devrait mener à une limitation très forte de la présence de microplastiques intentionnellement ajoutés dans différents produits, comme dans les granulats. Ces avancées très concrètes sont soutenues par la France.

en particulier en lien avec les émissions de composés volatils. » Finalement, vous en arrivez à la conclusion qu'il faut poursuivre le travail et aider les élus. Je vous en remercie.

même si le Gouvernement semble avoir à coeur de s'engager pour la sauvegarde de notre patrimoine, il apparaît néanmoins qu'il reste des domaines dans lesquels les actes ne sont pas à la hauteur des attentes. Ce manque de considération à l'égard de notre patrimoine le conduit tout droit à sa stricte disparition. Pire, cette cette politique engendre la destruction volontaire de bon nombre de monuments historiques qui font la fierté, l'honneur et l'histoire de nos territoires. Je pense particulièrement à la destruction de moulins à eau qui datent parfois du Moyen Âge, comme c'est le cas dans mon département de l'Orne. Outre que cette politique de continuité écologique sur la libre circulation des sédiments conduit à la démolition pure et simple de notre patrimoine, sa mise en oeuvre, sous ses aspects « écologiques », est en réalité désastreuse pour la sauvegarde et la protection des zones humides, souvent mal inventoriées, mais véritables viviers de la faune et de la flore dans nos territoires. Ce sont en effet des milliers d'écosystèmes à l'équilibre trouvé depuis plus de deux siècles qui se retrouvent menacés par ces destructions indirectes de milieux sauvages qui entraînent des ruptures d'équilibres naturels. Au-delà du coût environnemental, la continuité écologique a aussi un coût financier. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable estime la somme annuelle à la charge de l'État, des collectivités et des exploitants à près de 2 milliards d'euros. Une France championne de la dépense publique, composée de collectivités locales dépouillées de leur autonomie financière, n'a pas les moyens de se le permettre. Enfin, cette politique met un frein considérable à la transition écologique. En effet, la destruction d'anciens édifices, au-delà de son impact financier, patrimonial et environnemental, entrave le développement de la microélectricité, engendrant l'absence de production d'électricité par les différents sites déjà destinés à cet effet pour une durée qui peut aller jusqu'à huit ans. La continuité écologique apparaît ainsi plus que contre-productive sur le plan écologique et environnemental, outrancière sur le plan économique et désastreuse sur le plan patrimonial. patrimonial. Quelle alternative à cette politique de continuité écologique plus respectueuse du patrimoine et de la biodiversité entendez-vous mettre en oeuvre ?

et la biodiversité. Cette importance a d'ailleurs été réaffirmée par les Assises de l'eau et a été inscrite dans le plan Biodiversité, qui prévoit de restaurer la continuité sur 50 000 kilomètres de cours d'eau d'ici à 2030.

en particulier. Une analyse de la dimension patrimoniale des ouvrages hydrauliques a été élaborée. Elle a été transmise aux services déconcentrés comme élément à compléter pour

apaisée de la restauration de la continuité. Dans ce cadre, une instruction du 30 avril 2019 demande aux services déconcentrés de mieux tenir compte de cette dimension dans les choix d'intervention sur les ouvrages. En aucun cas

En 2004, l'État avait décidé de conserver dans son giron les routes nationales 19 et 57 qui irriguent le département de la Haute-Saône, en raison de leur caractère structurant pour le territoire national. Depuis, la logique d'itinéraire de la RN57 a été cassée, avec un tronçon Luxeuil-les-Bains-Vesoul qui doit passer sous la compétence du département dès que la RN19 sera modernisée en 2x2 voies sur la totalité du tronçon entre l'A36 et Vesoul. la modernisation de la RN19 suscite de nouveau des inquiétudes. Celles-ci se sont d'ailleurs vérifiées pour le tronçon ouest entre Vesoul et Langres qui, selon la lettre que Mme Borne m'a adressée le 9 mai 2019, ne fera plus l'objet que de travaux de déviations de villages et de sécurisations de carrefours.

et les différentes collectivités. Il est prévu que les préfets soient mandatés pour organiser cette concertation. Le réseau routier national non concédé fait bien sûr partie des compétences qu'il conviendra d'examiner et je peux vous assurer que le département de la Haute-Saône sera bien évidemment consulté. Je sais, monsieur le sénateur, que vous serez très vigilant sur cette question. L'État n'est pas fermé aux propositions des collectivités de faire évoluer leur implication dans sa gestion du réseau routier national, bien au contraire. C'est ce que montre l'adoption de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. Cette loi prévoit le transfert au 1 janvier 2021 de la totalité du réseau routier national non concédé à la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) et à l'Eurométropole de Strasbourg. Ce transfert couvre également le réseau autoroutier non concédé- l'A35 et l'A36 -, qui est transféré sous statut autoroutier Vous m'interrogez enfin sur les modalités de mise en oeuvre d'une décentralisation de certains axes du réseau routier national. Je souligne à nouveau l'intérêt de la loi du 2 août 2019 qui fixe pour la CEA les conditions auxquelles l'État va transférer le réseau routier national, tant sur le plan financier que sur celui des moyens. Il conviendrait de reconduire un tel dispositif lors d'un nouveau transfert de certaines routes nationales pour les collectivités qui se déclareraient intéressées. Voilà, monsieur le sénateur, notre volonté d'aller de l'avant sur l'importante question que vous soulevez.

D'abord, chez soi, il faut trouver la station-service : 6 pour les 6 000 routes du département de l'Aveyron, toutes avec des ouvertures programmées en journée, pause de midi comprise, et une seule accessible 24 heures sur 24 pour tout le département. Ensuite, il faut dénicher la pompe, installée souvent dans des endroits improbables de la station-service. Ailleurs, dans des secteurs plus fournis en autoroutes que l'Aveyron, tout semble de prime abord plus facile. Les stations affichent pour la plupart le GPL, mais il faut alors compter sur les pannes, les abandons du service sans explication, les réparations du matériel de distribution ... Mon collègue Jean-Claude Luche veut bien croire que le GPL porte encore la lourde charge d'être une énergie fossile et que les mesures de sécurité imposent des normes. il considère, à l'heure de la transition écologique chère au Gouvernement, que la mise à disposition de ce carburant relève de la discrimination. L'automobiliste GPL teste en grandeur nature ce que pourrait être demain la circulation avec des voitures électriques si l'on ne tient pas compte de la leçon : chaotique

de ce carburant ont été divisées par deux. Le GPL est le carburant alternatif qui bénéficie aujourd'hui du maillage le plus dense, capable d'assurer l'approvisionnement d'un parc de véhicules dix fois supérieur au parc roulant

issu principalement du raffinage des huiles végétales ou de production de bio-isobutène à partir de sucres, pourrait contribuer à renforcer l'attractivité de la filière et donc son développement, qui participe pleinement de la lutte contre les émissions de CO2. La parole

la taxe sur les passagers maritimes embarqués (TPM) est prévue par l'article 285 du code des douanes et est perçue lors de l'embarquement de passagers à destination des espaces protégés mentionnés à l'article D. 321-15 du code de l'environnement. Ce dernier mentionne donc la liste des espaces protégés et des ports les desservant, ainsi que la part du produit de la taxe et la personne publique bénéficiaire. Les falaises nord-est de Marie-Galante en Guadeloupe font partie des sites protégés mentionnés par ledit article dans le code de l'environnement. Afin que la communauté de communes de Marie-Galante puisse bénéficier de cette taxe, il conviendrait que la mention de l'ensemble des ports de Marie-Galante figure dans la liste de l'article D. 321-15 du code de l'environnement, ce qui permettrait l'assujettissement à la TPM, ainsi que l'a préconisé le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics lors de sa réponse à la présidente de la communauté de communes de Marie-Galante dans son courrier du 17 avril 2019. Ainsi, madame la secrétaire d'État, je vous demande de bien vouloir préciser dans quelle mesure le décret n° 2014-1197 du 17 octobre 2014 sera modifié afin d'y ajouter l'ensemble des ports de Marie-Galante.

en application de l'article D. 321-15 du code de l'environnement, la taxe prévue à l'article 285 du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime, dite taxe Barnier », est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement. Elle est perçue par la personne publique qui assure la gestion de l'espace protégé et est affectée exclusivement à la préservation de celui-ci. nous demandez, monsieur le sénateur, de vous préciser dans quelle mesure le décret n° 2014-1197 du 17 octobre 2014 pourrait être modifié de façon à prévoir que la taxe prélevée sur les entreprises chargées d'organiser le transport maritime de passagers vers le site classé des falaises nord-est de Marie-Galante soit effectivement perçue perçue par la communauté de communes de Marie-Galante. Sur la base de votre saisine, monsieur le sénateur, j'ai demandé aux services du ministère de la transition écologique et solidaire d'évaluer, en liaison avec les services de l'État en Guadeloupe, les modalités d'une éventuelle inscription de l'ensemble des ports de Marie-Galante sur la liste figurant à l'article D. 321-15 du code de l'environnement. Nous avons bien entendu votre requête et nous vous tiendrons au courant

Votre question renvoie aux multiples inquiétudes suscitées, à juste titre, par l'état de notre réseau ferroviaire de desserte fine du territoire, sur lequel les limitations de vitesse se multiplient. Comme cela a pu être rappelé à de nombreuses reprises par le Gouvernement ces derniers mois, les besoins nécessaires pour remettre à niveau ces lignes, si importantes pour la vitalité de nos territoires, pour les connexions locales, s'élèvent à plusieurs centaines de millions d'euros par an pour les dix prochaines années. Je vous confirme que l'État demeurera aux côtés des collectivités territoriales pour préserver ces lignes dans tous les territoires où ce mode de transport trouve encore sa pertinence et pour définir une priorisation des actions à entreprendre. Les défis étant nombreux, il nous faut donc prioriser.

7 millions d'euros en 2019 au titre du contrat de plan État-région 2015-2020 de la région Occitanie, ce qui a permis à l'ensemble des partenaires de signer la convention de financement des travaux programmés Ces travaux compléteront notamment ceux qui ont été réalisés au printemps 2019 sur la partie limousine de la ligne entre Brive et Saint-Denis-près-Martel, pour lesquels l'État a apporté 2 millions d'euros en 2017 au titre du contrat de plan État-région 2015-2020 de la région Nouvelle-Aquitaine. Dans son discours du 1 octobre 2019, le Premier ministre a confirmé qu'il convenait de développer un « bouquet de solutions » adaptées à chaque situation, et qu'un travail partenarial avec les régions et SNCF Réseau sera lancé pour élaborer des plans d'action concrets ligne par ligne. Il nous faut aller aussi précisément que possible dans le détail du maillage territorial pour répondre aux besoins spécifiques de chaque territoire. En tout cas, monsieur le sénateur Delcros, je vous remercie de votre question. Je vais alerter

territoriales. Madame la ministre, dans son rapport remis au Premier ministre au sujet d'une possible fusion du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence,

d'exercer et d'assurer la compétence voirie au 31 décembre 2019. Je me réjouis donc de l'adoption par le Sénat voilà quelques jours d'un amendement ayant pour objet de Néanmoins- je le sais pour me déplacer souvent dans les communes -, les maires ne se contenteront pas d'un simple report ; ils souhaitent garder la compétence, et je les comprends. et proximité dont nous débattons actuellement au Sénat et de son intitulé, vous portez une attention particulière à la réactivité des pouvoirs publics et à leur proximité. Après l'eau et l'assainissement, le report de ce transfert de compétence, qui- j'en suis sûre -fera naître l'espoir d'un énième report, place les maires dans une situation délicate délicate dans la gestion financière de leur commune. Pouvez-vous nous en dire plus sur les intentions du Gouvernement concernant cette compétence ?

Madame la sénatrice, nous le savons tous, Marseille a besoin d'une métropole forte, tout comme l'aire métropolitaine de Marseille a besoin d'une ville-centre forte.

Elles sont les moteurs d'une « alliance des territoires », ainsi qu'un rempart contre les fractures territoriales. L'État a le devoir d'encourager la coopération pour que le dynamisme et la solidarité entre les territoires soient effectifs. Au cas présent, l'enjeu est de taille. Il s'agit de permettre à Marseille, cette très grande ville française, symbole de la Méditerranée, de répondre aux défis du présent et de l'avenir.

exercent de plein droit la compétence voirie sur l'ensemble des voies communales appartenant à leurs communes membres. Pour la métropole Aix-Marseille-Provence, le transfert de la compétence était prévu au 1 janvier 2016.

par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Le Gouvernement est conscient que les conditions ne sont pas réunies pour que le transfert de l'ensemble de la compétence voirie prévu par la loi se déroule dans

réponse. Comprenez que les maires sont loin d'être des entraves aux réformes ; ils en sont plutôt demandeurs. Néanmoins, la gestion quotidienne de leur commune « en bon père de famille » nécessite de la visibilité,

Ma question porte sur les contraintes fortes liées à l'application du règlement de défense incendie et secours dans le département de la Seine-Maritime, et plus généralement sur les lourdeurs des normes qui pèsent sur les communes. En application de la loi Warsmann du 17 mai 2011, dont l'objectif premier est la simplification du droit, le maire « assure la défense extérieure contre l'incendie ». Or, en Seine-Maritime, force est de constater que les modalités d'application du référentiel national d'incendie et de secours sont loin de simplifier la vie des maires À tel point que le préfet a dû s'y reprendre à deux fois pour élaborer le règlement départemental incendie et secours, finalement adopté le 26 octobre 2017. Depuis, sa mise en oeuvre crée toujours autant de difficultés, notamment dans les communes rurales. La sécurité des habitants est une priorité pour tous les maires. Mais l'interprétation souvent très stricte et peu pragmatique des dispositions de ce règlement départemental en Seine-Maritime génère des contraintes disproportionnées sur certains territoires. L'appréciation de la distance entre le point d'eau et l'habitation est en effet source de difficultés. Le règlement dispose que toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne à incendie ou à moins de 400 mètres si l'habitation est isolée. Ce principe d'interprétation très stricte a des conséquences désastreuses sur la capacité des communes à délivrer de nouveaux permis de construire. De même, l'interprétation du calibrage des réserves à incendie suscite de fortes incompréhensions chez les élus. Les maires, dépossédés de leurs prérogatives d'urbanisme au profit des intercommunalités, contraints en zone littorale par la protection des rivages et limités par l'application stricte du règlement départemental incendie et secours, n'ont plus aucune marge de manoeuvre pour l'aménagement du territoire communal.

Madame la sénatrice, chère Agnès Canayer, je vous prie d'excuser l'absence de M. le ministre de l'intérieur ; je répondrai à sa place. La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire

mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet. L'objectif est double : une concertation renforcée avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse pour des mesures adaptées à chaque territoire. Ce règlement est élaboré par le

Ses préconisations s'appuient sur des objectifs de sécurité et sur une analyse des risques répondant de la manière la plus adaptée à la diversité des risques au sein du département.

Dans le département de la Seine-Maritime, l'adoption du règlement de la DECI en février 2017 a suscité de nombreuses réactions de la part des élus. En conséquence, la préfecture l'a révisé en révisé en octobre 2017 après concertation avec les représentants des collectivités territoriales. Cette révision a recueilli le soutien des élus locaux. Par ailleurs, les communes ou les EPCI peuvent mettre en place un schéma communal ou intercommunal de DECI. Ce document permet notamment

s'agissant des compétences relevant des collectivités territoriales. Je rappelle que toutes les possibilités juridiques et techniques offertes dans le cadre de la DECI doivent être utilisées dans les territoires pour déployer des réponses réalistes et adaptées. Enfin, le ministère de l'intérieur n'élaborera pas de dispositions qui contraindraient le contenu des règlements départementaux. Cela serait évidemment en opposition avec les fondements mêmes de la réforme de 2015, déployés sur le terrain de 2016 à 2017. Il convient de laisser le temps nécessaire à cette mise en place et à la réalisation

qui fixe les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire dans l'attente de la réalisation de la crémation ou de l'inhumation définitive. Cet article autorise notamment le dépôt temporaire d'un cercueil dans des édifices « cultuels », définis comme des édifices « clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte ». En revanche, il interdit le dépôt « en dépositoire » sauf si le dépositoire est situé dans l'enceinte d'un cimetière, comme si un mur d'enceinte avait des propriétés sanitaires ... Il s'ensuit, notamment en Moselle, que les communes ne peuvent plus du tout utiliser leurs dépositoires, obligeant le plus souvent des personnes âgées, voire très âgées, et déjà durement éprouvées par la perte d'un être cher, à effectuer de longs et pénibles déplacements jusqu'à la morgue la plus proche,

de manière à rétablir la règle qui prévalait antérieurement. Y êtes-vous favorable ? la ministre. Monsieur le sénateur, conformément aux dispositions de l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, le corps des personnes décédées peut faire l'objet, après la mise en bière, d'un dépôt temporaire. Le dépôt temporaire du cercueil débute alors, dans la limite du délai légal d'inhumation, à savoir six jours au plus tard après le décès. Comme vous le rappelez très justement, la réglementation détermine de manière limitative les lieux où le dépôt temporaire des cercueils est autorisé. Ainsi, ce dépôt est autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt, voire à celle d'un membre de sa famille ou, enfin, dans un caveau provisoire. Dans la seule hypothèse du caveau provisoire, la durée autorisée de dépôt temporaire est alors non plus de six jours, mais de six mois, durée maximale et non renouvelable. Par ailleurs, et c'est sur ce point que vous attirez mon attention, l'article R. 2213-29 du CGCT a été modifié par le décret du 28 janvier 2011, afin d'y ôter toute référence au « dépositoire Les dépositoires étaient tantôt des équipements sous forme de cases séparées par des cloisons sommaires, tantôt des bâtiments pouvant contenir des cases destinées à accueillir les cercueils. Les dépositoires avaient ainsi la particularité d'être situés en surface. Tout comme les caveaux provisoires, ils étaient gérés par la commune. La suppression du terme « dépositoire » et par là même l'interdiction de leur utilisation avaient pour objectif d'éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d'assurer la sécurité sanitaire. Toutefois, dans la pratique, il demeure possible d'assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des caveaux provisoires, même lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs cases situées au-dessus du niveau du sol. Ainsi, les structures existantes, à condition qu'elles demeurent bien dans l'enceinte du cimetière communal, peuvent toujours être utilisées pour un dépôt temporaire. Elles correspondent juridiquement aux « caveaux provisoires », dont les modalités de gestion et d'utilisation doivent être détaillées dans le règlement du cimetière communal.

ma question porte sur les modalités d'institution, de renonciation et de suppression de la taxe d'aménagement par les communes ou EPCI. La communauté d'agglomération du Grand Besançon est passée en communauté urbaine le 1 juillet dernier. Ce changement de statut implique notamment que la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans la nouvelle collectivité. 3° de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme dispose que la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communautés urbaines sauf renonciation expresse décidée par délibération. Or il est difficile de déterminer si le troisième alinéa s'applique de manière exclusive ou non du deuxième du même article, qui est la possibilité pour une commune de prendre une délibération pour restituer cette taxe.

La communauté urbaine délibérera ce jeudi sur cette question. Elle s'est engagée à restituer ce que rapporterait la taxe aux communes. Or les maires sont inquiets et craignent que la part restituée ne s'amenuise d'année en année. C'est pourquoi plusieurs maires souhaiteraient que la communauté urbaine renonce à percevoir la taxe d'aménagement. Mais l'inconnue réside dans les conséquences de cette renonciation. Dans l'exposé de l'article 14 du projet de loi de finances rectificative pour 2010, qui a créé la taxe d'aménagement, il est indiqué que la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes urbaines et par délibération dans les autres communes. Cette formulation n'est pas dépourvue d'ambiguïté quant aux conséquences d'une renonciation par la communauté urbaine à l'institution de la taxe. L'intention du législateur n'apparaît pas clairement. Madame la ministre, pour ce qui est de la taxe d'aménagement, dans le cas où la communauté urbaine renoncerait expressément à instituer une part intercommunale, est-il possible pour les conseils municipaux d'instituer une part communale ? Je souhaiterais avoir un avis circonstancié permettant de fixer cette doctrine doctrine administrative. La parole est à Mme la ministre. Monsieur le sénateur, la taxe d'aménagement est composée de trois parts : la part communale ou intercommunale, selon l'autorité compétente pour l'instituer, la part départementale et, pour la seule région Île-de-France, la part régionale. L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme fixe les conditions d'institution de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement. Cette dernière est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. Dans les autres communes, elle peut être instituée par délibération du conseil municipal, et pour une période minimale de trois ans. Lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, ce dernier peut percevoir en lieu et place de la commune la part de la taxe d'aménagement qui lui revient ; la part communale devient alors alors intercommunale. Ainsi, les communautés urbaines et les métropoles en dehors de la métropole du Grand Paris sont compétentes de plein droit pour percevoir la part intercommunale. Dans les autres EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme, elle pourra être instituée pour une durée minimale de trois ans par délibération du conseil communautaire avec l'accord des communes membres exprimé à la majorité qualifiée.

en matière de taxe d'aménagement. Si une commune ou un EPCI compétents de plein droit pour percevoir la part communale ou intercommunale ne souhaitent pas percevoir le produit de cette part, ils peuvent y renoncer par délibération. Cette délibération devra être prise avant le 30 novembre pour entrer en vigueur chaque année le 1 janvier. Elle est valable, selon les termes du dixième alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur. il ne sera plus perçu de part communale ou intercommunale pendant la durée de la validité de la délibération de renonciation. La renonciation à percevoir le produit de la taxe par un EPCI n'a pas pour effet de transférer la possibilité d'instituer une part communale aux communes. En effet, le code de l'urbanisme ne prévoit pas le transfert de cette compétence de plein droit, acquise par la loi, par la communauté urbaine ou la métropole à ses communes membres, qu'il y ait renonciation ou non par cette collectivité. En revanche, les communes membres des EPCI non compétents de plein droit en matière de taxe d'aménagement et devenus compétents par délibération des communes peuvent décider à la majorité qualifiée et à l'issue de la période minimale d'instauration de trois ans de récupérer cette compétence. Enfin, afin de tenir compte de la charge que le coût des équipements publics fait peser sur les budgets des collectivités, lesquelles ne sont pas nécessairement celles qui perçoivent la taxe d'aménagement, il y a un alinéa qui prévoit un mécanisme de reversement de la part intercommunale aux communes. Dans ce cas, l'EPCI pourra prendre à tout moment une délibération fixant les conditions de reversement de tout ou partie de la part intercommunale à ses communes membres.

sans doute que le Gouvernement va mettre en place des maisons France services pour remplacer les structures ainsi supprimées. Beaucoup d'élus redoutent que la qualité de service ne soit pas la même

Le Président de la République et le Premier ministre ont réaffirmé leur attachement à la proximité en matière de services publics. M. le Premier ministre déclarait ici même le 13 juin vouloir « reconstruire un vrai maillage cohérent de présence des services publics ».

par semaine, dans lequel il pourra obtenir des réponses complètes sans réorientation systématique à des démarches du quotidien. France services repose avant tout sur une exigence de qualité.

de la formation proposée aux agents polyvalents pour que chacun puisse être pleinement informé des démarches propres à chacun des neufs partenaires-socles du bouquet de services Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, La Poste, la DGFiP, le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur. Chaque agent bénéficiera avant toute ouverture d'une maison France services de cinq jours et demi de formation en présentiel tant sur la partie « socle commun posture de l'agent, médiation numérique et maîtrise des outils numériques de la maison -que sur la partie « métier », c'est-à-dire des modules organisés par situation de vie dispensés par des formateurs de chacun des neuf partenaires du bouquet de services. J'insiste ce point, car la formation des personnels est très importante. Une relation privilégiée sera garantie entre les agents polyvalents des maisons et leurs interlocuteurs locaux désignés dans chacune des neuf structures partenaires. Les outils informatiques développés par la direction informatique de l'État et la Banque des territoires faciliteront la tâche de ces agents dans la résolution des requêtes plus ou moins complexes. Il y aura aussi des organisations de visioconférence dans un espace de confidentialité de confidentialité prévu à cet effet. Les premières structures France services seront labellisées au début de l'année 2020. Bien évidemment, il s'agit de labelliser soit des maisons qui existent déjà et qui sont au niveau, soit des créations nouvelles. Dans le

il peut y en avoir trois ou quatre par canton.

Madame la ministre, je souhaite interroger le Gouvernement sur les difficultés récurrentes rencontrées par nos concitoyens qui souhaitent faire construire et s'installer en milieu rural, dans des secteurs le plus souvent à très faible densité de population. En effet, trop souvent, ceux-ci se voient opposer un refus par les services de l'État, qui ne connaissent évidemment pas précisément le site concerné, alors même que celui-ci est en prise directe avec tous les réseaux de viabilisation et qu'il n'y a sur le aucune pression foncière agricole, et au seul motif que la parcelle concernée n'appartiendrait pas- le terme est succulent -à un « compartiment

totalement antinomiques avec le discours ambiant que vous portez à bon droit sur la cohésion des territoires, mais qui demande des traductions locales. Ces élus nous interpellent régulièrement. Il leur arrive en dernier recours de saisir personnellement le préfet, qui peut procéder au cas par cas à une application plus souple, voire plus intelligente de la loi et des règlements

intercommunal (PLUI) ou de documents d'urbanisme, dans la partie déjà urbanisée d'une commune, conformément au règlement national d'urbanisme. Ce principe vise à inciter les collectivités à organiser la gestion de leur sol et à lutter sol et à lutter contre l'urbanisation dispersée, en autorisant toutefois certaines exceptions, comme les constructions de logements, notamment pour le maintien de la population communale dès lors qu'une délibération motivée du conseil municipal est prise en ce sens. Autrement, les territoires ruraux peuvent choisir de se doter d'un plan local d'urbanisme, communal ou intercommunal, pour définir une capacité de construction et d'ouverture à l'urbanisation supplémentaire, notamment au regard d'un diagnostic foncier de capacité de desserte en voirie et réseaux, mais aussi pour pouvoir construire sous certaines conditions, dans des zones agricoles ou naturelles, dans des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées. Ainsi, sur la période 2006-2014, on a pu observer que dans les zones rurales, avec une augmentation de 3 % des ménages, la consommation des espaces a représenté

de pouvoir développer l'urbanisation et l'habitat ainsi que la volonté de lutter contre l'usage d'une ressource non renouvelable qu'est le sol. Je partage votre souci de réduire les inégalités territoriales et de maintenir l'attractivité du territoire. C'est en ce sens que j'ai, conjointement avec Didier Guillaume, installé une mission pour identifier et prioriser les mesures de soutien au développement des territoires ruraux en matière d'urbanisme dans le cadre de l'Agenda rural. La mission plaide ainsi pour un meilleur accompagnement des collectivités, notamment

sur le fait que l'une des entreprises chargées du chantier de la gare d'Austerlitz à Paris a été conduite à interrompre ses travaux en raison de taux de plomb, qui, selon elle, étaient alarmants

Cela a suscité des réactions compréhensibles de la part des syndicats de personnels de la SNCF, des entreprises qui travaillent sur ce vaste chantier,

été relevé. La gare de Paris-Austerlitz fait en effet l'objet d'importants travaux de modernisation. Ils concernent notamment la rénovation complète de la Grande halle voyageurs, qui comprend un décapage complet des charpentes métalliques, historiquement peintes avec des peintures au plomb, peintures au plomb, et la dépose des éléments en bois, eux-mêmes souvent peints avec ce type de peinture. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France est, depuis le début du chantier, mobilisée sur le sujet. Des investigations sont en cours pour apprécier l'impact sanitaire de cette pollution au plomb sur la population générale éventuellement exposée dans la gare ou aux abords immédiats de celle-ci. Les travaux sont menés sous confinement, afin que les particules de plomb tombant au sol dans la zone du chantier ne puissent s'en échapper. Ils font par ailleurs l'objet d'un suivi particulier, avec notamment des relevés hebdomadaires de la de la présence éventuelle de plomb par un bureau d'études spécialisé. Les contrôles sont effectués dans l'ensemble de la gare et du chantier, y compris dans les zones accessibles au public. Depuis septembre 2018, sur l'ensemble des mesures réalisées, six valeurs ont été supérieures à 1 000 microgrammes par mètre carré, les dernières mesures effectuées début octobre dans les zones accessibles au public étant toutes inférieures à ce seuil. Cette valeur est prévue par l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb ; elle doit être respectée lors des contrôles réalisés en fin de travaux d'urgence visant à supprimer le risque d'exposition au plomb. Ce seuil traduit l'efficacité du nettoyage réalisé à la suite de travaux de suppression de l'accessibilité du plomb et les poussières retrouvées de manière résiduelle sont destinées, à terme, à disparaître. S'agissant particulièrement de la zone de chantier, des prélèvements ont constaté des niveaux supérieurs au seuil de 1 000 microgrammes par mètre carré, sans pour autant que ces niveaux atteignent la valeur limite d'exposition professionnelle réglementaire applicable aux travailleurs.

Cette réunion a permis de faire l'inventaire des mesures d'empoussièrement réalisées à l'initiative des différentes parties prenantes et de constater plusieurs irrégularités relatives aux zones de décontamination présentes. L'inspection du travail a donc demandé des mesures correctives adaptées aux différents intervenants. Le plan d'action de la SNCF doit être présenté rapidement au service de l'inspection du travail. Je suis

et de la santé. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite vous interroger au sujet de la démarche dite du « patient blood management » (PBM), autrement dit la gestion personnalisée du capital sanguin. J'associe à cette question mes collègues Corinne Imbert, Martine Berthet, René-Paul Savary et Jean Sol, puisqu'elle fait suite à une audition commune L'anémie préopératoire, le plus souvent causée par une carence martiale, est fréquente et constitue un facteur de risque d'augmentation des complications postopératoires. Pour y remédier, le traitement de première intention est le recours à la transfusion de concentrés de globules rouges. Les transfusions sanguines sont irremplaçables et sauvent des vies, mais les produits sanguins sont rares et précieux, chers et exposés à des risques de pénurie. L'enjeu est donc de gérer l'anémie au mieux tout en épargnant au maximum le recours à la transfusion sanguine, et d'utiliser la transfusion non plus comme le traitement par défaut, mais comme un ultime Pour y parvenir, le PBM vise à mettre en place une stratégie coordonnée, multimodale et multidisciplinaire, voire pluriprofessionnelle, fondée sur des concepts scientifiquement validés et centrés sur le patient. L'objectif est de maintenir des concentrations acceptables d'hémoglobine, d'optimiser l'hémostase et de minimiser les pertes sanguines. Cette démarche est recommandée par l'OMS, la Commission européenne et les sociétés savantes internationales. La Société française d'anesthésie-réanimation souligne la nécessité

La France accuse un retard manifeste et en est au stade de l'expérimentation. Si j'interviens ce matin, c'est parce que cette démarche a fait l'objet d'une expérimentation dans mon département, plus précisément au CHU d'Angers, sous la conduite du professeur Lasocki. Il s'agissait d'un programme « objectif zéro transfusion », qui incluait des patients admis pour une prothèse de hanche ou de genou. Les résultats cliniques ont été significatifs : augmentation des prescriptions justifiées d'EPO en préopératoire et de Fer IV et une nette baisse des patients transfusés. Depuis la mise en oeuvre du programme, le secteur anesthésie a diminué ses dépenses en produits sanguins de plus de 20 %. En conclusion, cette approche permet de diminuer considérablement le recours aux transfusions, les complications, la durée des séjours hospitaliers, la mortalité et les coûts.

et l'autosuffisance sont aujourd'hui assurés grâce au geste altruiste des donneurs et au professionnalisme de l'Établissement français du sang. La gestion personnalisée La gestion personnalisée du capital sanguin est une approche thérapeutique multidisciplinaire centrée sur le patient, visant à optimiser la prise en charge dans un contexte transfusionnel. Agnès Buzyn y est donc particulièrement sensible, comme à toute démarche favorisant la qualité et la pertinence des soins pour le patient. patient. La définition d'une politique de transfusion sûre et rationnelle favorisant, chaque fois que possible, des mesures d'épargne sanguine fait déjà l'objet de recommandations professionnelles. Mais il est vrai que cette approche,

D'une part, pour évaluer et favoriser le déploiement de ces bonnes pratiques médicales et organisationnelles, la Haute Autorité de santé sera sollicitée afin de compléter ses recommandations sur la transfusion sanguine s'intégrant dans le cadre de la récupération améliorée après chirurgie (RAAC) et, le cas échéant, afin d'intégrer les enjeux des protocoles de gestion personnalisée du capital sanguin en pré, per et postopératoire. Les sociétés savantes vont réaliser en 2020 une étude sur les données collectées dans le cadre des expériences actuellement menées dans 15 établissements de santé. Ces résultats permettront d'objectiver, à partir d'indicateurs, l'amélioration de la qualité de prise en charge des patients et le gain médico-économique associé à cette démarche. D'autre part, plusieurs mesures d'accompagnement du développement de la chirurgie ambulatoire et de la réduction des durées de séjours chirurgicaux ont été mises en place lors de la campagne tarifaire 2019. En particulier, un soutien au développement de l'activité de RAAC, qui inclut la gestion de l'anémie préopératoire, est d'ores et déjà mis en oeuvre depuis mars 2019.

Les médecins souhaitant devenir maîtres de stage universitaire doivent adresser leur demande auprès du département de médecine générale le plus proche et dans la même région que celle du lieu d'exercice de leur activité.

voisins de l'UFR de Saint-Quentin-en-Yvelines, la distance, qui s'ajoute aux nombreuses contraintes liées à leur profession, est un frein véritable à leur aspiration d'accueillir des étudiants. Et, pour le territoire, ce sont autant d'opportunités en moins de découvrir de nouvelles vocations au service d'un département parmi les plus déficitaires en médecine générale. Ainsi, et parce que ces rigidités administratives paraissent excessives dès lors que l'exercice de la profession est encadré par une inscription au tableau de l'ordre et un numéro d'identification des professionnels, je souhaiterais savoir s'il serait possible, dans la limite des capacités d'accueil, de déroger à ce principe pour permettre aux médecins souhaitant devenir maîtres de stage de s'inscrire dans le département de médecine générale et de suivre leur formation dans l'UFR le plus proche de leur lieu d'exercice, même si ces formations sont dispensées dans une autre région que celle où ils exercent leur activité.

pour permettre aux étudiants, futurs médecins, de se former et de découvrir un large spectre de situations professionnelles. C'est ainsi que pourront naître de nouvelles vocations, notamment dans des environnements plus éloignés ou différents des centres hospitaliers habituellement fréquentés, compte tenu des représentations que les futurs médecins pouvaient se faire eux-mêmes de leur propre profession. L'article 4 de la loi du 24 juillet 2019 prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les règles d'agrément des praticiens maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité ». Une concertation associant l'ensemble des parties prenantes vient d'être lancée afin d'améliorer et de faciliter le processus d'accès à la maîtrise de stage des praticiens. Cette concertation permettra d'alimenter le projet de décret dont la finalisation est attendue pour le début de l'année 2020. La liberté de choix de l'université ou de l'organisme formateur sera réaffirmée dans ce décret.

En Picardie, le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide en médecine-chirurgie, chez les jeunes filles de 10 à 14 ans, s'élève à 7,3 pour 10 000 habitants. Chez les jeunes filles de 15 à 19 ans, il est de 90 pour 10 000 habitants.

Hélas, le département ne possède aucun sociologue ni aucun service permettant de faire des relevés de statistiques et d'analyses précis sur ces deux thématiques. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais les facteurs de vulnérabilité des jeunes s'accentuent avec la précarisation et la dégradation du niveau socioculturel de la population. En 2009, 8,3 % des jeunes

Le taux de pauvreté est aussi largement supérieur à la moyenne nationale. Monsieur le secrétaire d'État, l'Aisne ne dispose d'aucun outil adapté pour répondre à cette problématique des adolescents et adolescentes. Les soignants de l'établissement de santé mentale du département de l'Aisne, très actifs, proposent la mise en place d'un groupe de recherche et de réflexion avec l'ensemble des partenaires et des services publics concernés.

qui concernent à la fois le repérage et l'orientation pour les citoyens ou les professionnels non cliniciens. Le dispositif de recontact des suicidants « VigilanS est opérationnel depuis février 2019 sur les deux secteurs de psychiatrie gérés par le centre hospitalier de Saint-Quentin. Les jeunes patientes qui se présenteraient ainsi dans cet établissement peuvent bénéficier du dispositif, tout en étant suivies parallèlement en pédopsychiatrie. Par ailleurs, l'installation d'une maison des adolescents dans l'Aisne en 2020 est à l'étude, avec un portage confié à la ville de Saint-Quentin. L'IVG et les grossesses chez les jeunes filles de moins de 16 ans font l'objet d'une attention toute particulière des autorités sanitaires, même s'il s'agit d'événements rares,

a également développé une application mobile, « Bien dans ma sexualité », qui permet de valoriser l'offre en santé sexuelle et de la rendre accessible. Disponible dans toute la région, elle a été téléchargée près de 400 fois depuis décembre 2018. Enfin, des projets ont été déployés dans le cadre du parcours éducatif de santé, en liaison avec l'éducation nationale. Le projet de prévention par les pairs développé par le collège de Vic-sur-Aisne en est un bon exemple. Le

fermeture des services de néonatalité, réanimation et pédiatrie, menaçant en outre les services de maternité et de chirurgie, programmation de la suppression de 90 lits et de 200 postes de travail. Les choses sont arrivées à échéance en septembre de cette année. « Mme la maire de Méru, M. le maire de Chantilly et M. le maire de Butry avaient demandé que ces mesures soient abandonnées et que vous puissiez les recevoir.

L'objectif de cette réorganisation est de parvenir à maintenir une activité de médecine, chirurgie ambulatoire et obstétrique sur le site de Beaumont-sur-Oise, le plus impacté par ces difficultés, en favorisant notamment le développement de l'activité de maternité. Il ne s'agit ni de fermetures de services ni d'une fermeture de lits disséminée sur l'ensemble du département, encore moins de fermetures d'hôpitaux, mais de la mise en place d'équipes territoriales, mutualisées

Par ailleurs, le projet de reconstruction de l'hôpital d'Argenteuil a récemment été jugé éligible par le Comité interministériel de validation des projets d'investissement, le Copermo, et devrait donc pouvoir être enclenché dans les mois à venir. La

à des analyses de la terre qui les entoure. Les résultats seraient particulièrement alarmants. Des parents s'interrogent par ailleurs : pourquoi limiter aux enfants de moins de 11 ans la surveillance clinique et biologique individuelle à l'exposition à l'arsenic

Les pouvoirs publics ont certes pris nombre d'initiatives, mais, au vu des résultats des analyses et des indications diverses qui nous parviennent, il faut donner un signal fort à la population. L'urgence le commande ! Il est donc impératif qu'une enquête épidémiologique soit engagée pour toute la population. Un plan de prélèvement est-il envisagé, monsieur le ministre, afin de mesurer les conséquences à terme sur les populations exposées ? Je suggère par ailleurs l'installation d'un centre de suivi médical

Enfin, pour éviter que, lors de prochaines intempéries, les mêmes causes ne produisent les mêmes effets en matière de pollution, quand va-t-on se débarrasser de cette montagne de déchets du site de Nartaud, qui stocke 85 000 tonnes

initiales de l'Agence régionale de santé (ARS) ont été complétées par une notice d'information, un dossier de questions-réponses relatif à la situation sanitaire de ce site et un dispositif téléphonique et de messagerie pour répondre aux questions de la population.

réalise, quant à elle, une nouvelle campagne d'analyse d'échantillons de légumes issus des jardins potagers inondés en vue d'évaluer leur éventuelle contamination. En termes de surveillance sanitaire des populations, l'ARS a saisi Santé publique France en mai pour évaluer le risque sanitaire actuel et la pertinence de réaliser de nouvelles études épidémiologiques ou d'actualiser celles qui ont déjà été réalisées. En termes de surveillance sanitaire individuelle, la direction générale de la santé a saisi la Haute Autorité de santé afin qu'elle établisse en partenariat avec la Société de toxicologie clinique des recommandations concernant le dépistage, le suivi et la prise en charge des personnes potentiellement surexposées à l'arsenic du fait de leur lieu de résidence.

et des femmes enceintes, populations particulièrement vulnérables, vous en conviendrez. Et les autres ? Ce dispositif a été mis en place à partir du 8 juillet 2019 en liaison avec les professionnels de santé de la vallée de l'Orbiel et le Centre antipoison et de toxicovigilance de la région Occitanie. L'ARS prend à sa charge le financement de ces analyses biologiques. Les consultations médicales et les éventuels examens complémentaires sont pris en charge suivant les modalités usuelles par l'assurance maladie- sécurité sociale et mutuelles. Un communiqué de presse conjoint de la préfecture de l'Aude et de l'ARS du 7 octobre 2019 octobre 2019 indique que les résultats des études du BRGM et leur analyse par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) ont été transmis à Santé publique France dans le cadre de la saisine de l'ARS sur la pertinence de mener d'autres études de santé. Les deux rapports de l'Ineris sont accessibles sur les sites internet de la préfecture de l'Aude et de l'ARS. Les résultats du dispositif de suivi médical mis en place pour les enfants de la vallée de l'Orbiel sont en outre mis à jour régulièrement sur le site de l'ARS-

à savoir une surmortalité préoccupante dans l'agglomération nazairienne. En effet, il existe une surmortalité de 28 % chez les moins de 65 ans, 41 % de celle-ci étant due à des cancers, 30 % de ces derniers étant prématurés chez les hommes, 12 % chez les femmes.

Se côtoient dans ce secteur différentes industries telles que la construction navale, l'aéronautique ou les industries chimiques et pétrolières, autour d'un grand port maritime. Est-ce la conjonction de ces éléments, notamment les rejets de ces activités dans C'est pourquoi une enquête épidémiologique de grande envergure est indispensable pour en connaître précisément les origines, ainsi qu'une étude beaucoup plus récente sur les causes de mortalité. Pour cela, il est nécessaire que des crédits de recherche spécifiques soient débloqués urgemment sur la problématique liée à ce secteur géographique, car personne ne pourra accepter une telle inégalité territoriale d'espérance de vie. Par ailleurs, un suivi permanent de l'évolution des constats et des décisions prises sera indispensable. Les élus, les responsables économiques et le tissu associatif attaché à cette problématique de santé devront être régulièrement informés des évolutions constatées et des orientations qui auront été décidées. La transparence, monsieur le ministre, est primordiale afin d'alerter, sans paniquer, d'informer avec objectivité et d'appréhender les éléments de prévention. Je compte sur vous pour prendre en considération ces différentes demandes afin de tirer véritablement les enseignements des résultats angoissants constatés par l'Agence régionale de santé sur l'agglomération nazairienne. La parole Yannick Vaugrenard, je ne peux que vous rejoindre sur l'impératif de transparence, d'autant plus quand la santé de nos concitoyens est en question. Vous l'avez souligné,

montrent une amélioration globale de la santé au sein de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (Carene), notamment en termes d'espérance de vie. Cette évolution demeure toutefois moins favorable qu'au niveau national. Les causes de cet état de santé globalement défavorable sont complexes à appréhender. De multiples facteurs, qui se cumulent et interagissent tout au long de la vie, peuvent être en cause, notamment des facteurs génétiques, liés aux comportements et habitudes de vie, aux expositions professionnelles et environnementales.

Sans attendre les résultats de ces nouvelles études, l'ARS et plusieurs communes de la Carene travaillent d'ores et déjà à un nouveau contrat local de santé qui, en 2020, pourrait s'élargir à l'ensemble du bassin nazairien. Les mesures de ce nouveau contrat local interviendront en complément des actions déjà entreprises dans le cadre du contrat en cours depuis 2015. Enfin, des

avec comme principale explication l'absence de rentabilité de cette technologie. En France, ces pompes sont utilisées par 250 patients diabétiques. À la suite de cette annonce, ces patients se sont vu proposer comme alternative une pompe externe ou un autre traitement. Malheureusement, pour 90 % d'entre eux, ces alternatives ne sont pas adaptées à leur pathologie. En effet, cette forme de diabète instable et ingérable nécessite un traitement très spécifique qui n'était jusqu'alors proposé que par l'entreprise Medtronic.

le ministère des solidarités et de la santé suit ce dossier avec une attention particulière. Des actions sont prises, à la suite de la réunion organisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en septembre dernier avec l'ensemble des parties prenantes, dont le collectif de patients concernés,

d'une part, veiller aux engagements pris par cette firme de garantir la disponibilité des consommables nécessaires au bon fonctionnement de ces pompes pour les patients utilisateurs, et, d'autre part, faire un point régulier sur les alternatives potentielles pérennes pour la fabrication de ces pompes.